M. Guillaume Gontard. Nous avons vu hier soir que cet article 22 posait problème. Les amendements de suppression n'ont pas été votés, mais on voit bien que la commission s'est posé des questions et a essayé d'encadrer l'usage des drones. Cet amendement, inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza, a justement pour objet de préciser et de renforcer la rédaction de l'actuel alinéa 6 pour garantir qu'en aucune façon des images de drones filmant l'intérieur des domiciles ne puissent être visionnées, comme le prévoit actuellement le texte. à compléter le dispositif en y ajoutant les espaces extérieurs privés et l'intérieur des véhicules. Le respect de la vie privée et de l'intimité des personnes doit être le même dans tous les cas, que l'on soit allongé sur son canapé, affairé dans son jardin ou au volant de sa voiture.

de manière à éviter toute ambiguïté concernant le champ visuel sur lequel les caméras aéroportées peuvent intervenir. Cette proposition rejoint donc la préoccupation de protection de la vie privée et du domicile.

Cette proposition de loi doit garantir une meilleure protection des forces de l'ordre et une plus grande efficacité de leurs actions sans tomber dans la tentation de Big Brother. Ces excès entraveraient les efforts légitimes qu'il est urgent et nécessaire de Il convient donc de refuser la reconnaissance faciale par les drones ou l'intrusion dans la vie privée des domiciles, et de l'écrire clairement dans cet article. Je souhaite cependant, par cet amendement, rétablir la possibilité pour les forces de l'ordre de filmer les parties communes des immeubles, qui sont des parties non privatives, ainsi que des entrepôts. Il n'aura échappé à personne que les halls d'immeubles sont souvent le lieu de nombreux trafics, en particulier des trafics de drogue, dans un grand nombre de cités marseillaises notamment. du regard des forces de l'ordre, et toujours au détriment des habitants des immeubles concernés, qui finissent par être pris en otage dans leur propre domicile. Il est également de notoriété publique que le mode de fonctionnement des Black Blocs ou autres mouvements d'extrême gauche

En effet, les halls d'immeubles servent à échapper aux fouilles des forces de l'ordre aux points d'entrée des manifestations et à y cacher du matériel qui deviendra ensuite des armes par destination. Ils servent également de refuge lorsque les forces de l'ordre tentent de procéder à des interpellations. Il paraît donc proportionné, pour le bien de tous, sans entrave à la vie et à la propriété privées, de permettre aux drones de capter des images dans les parties communes d'immeubles d'habitation ou d'entrepôts, dans le respect strict des dispositions de cet article.

on peut imaginer que les opérations de police aient besoin d'images captées depuis la voie publique dans des espaces qui, eux, ne sont pas ouverts au public, par exemple des parkings privés ou des entrepôts.

Je vais retirer l'amendement déposé par Hervé Marseille. Je pense que j'arriverai à le convaincre de la sagesse et de la pertinence des arguments du rapporteur et du ministre-

autant de lignes directrices permettant de préciser les exigences de formation des personnels, les garanties juridiques générales énoncées par la loi, les cas concrets où l'usage des drones peut être considéré comme proportionné au regard des finalités autorisées par la loi- c'est très important pour éviter les risques constitutionnels -, et surtout de définir les spécifications techniques qui, si elles n'ont pas leur place dans la loi,

le ministre, ainsi qu'au préfet de police de Paris, un véritable camouflet en interdisant d'utiliser les drones pour surveiller les rassemblements sur la voie publique. Dans sa décision, le Conseil d'État dénonçait même le dispositif dans son essence : « Le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement, dans les circonstances actuelles, en l'absence de recours à des drones. En droit des données personnelles, si l'utilité d'un dispositif de surveillance n'est pas clairement démontrée, celui-ci ne peut jamais être autorisé. Là où sont en cause des données sensibles telles que les opinions politiques captées en manifestation, il faut même, pour qu'ils soient autorisés, que ces dispositifs soient absolument nécessaires au maintien de l'ordre. Cette proposition de loi ne justifie en rien cette absolue nécessité. Rien ne vient donc justifier cette atteinte gravissime au droit de manifester et à la liberté d'opinion- nous en avons déjà parlé hier soir. Quel

en exigeant que des circonstances particulières soient réunies : lorsqu'il existe des craintes de troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, lorsque les circonstances liées au lieu de l'opération rendent difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou lorsque ces circonstances sont susceptibles d'exposer les agents à un danger significatif. Avec le dispositif proposé, nous pensons avoir bien encadré le problème. Avis défavorable.

à M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet l'utilisation des drones pour la surveillance des frontières. Je ne m'étendrai pas sur la politique migratoire de la France, aussi inhumaine qu'inefficace. Mais je vais tenter de vous convaincre avec des arguments rationnels. Le retour d'expérience de la surveillance de la frontière américano-mexicaine par drones fait état d'une immense gabegie financière : cette politique est coûteuse et inefficace. En 2015, un rapport du département de la sécurité intérieure faisait apparaître que les arrestations d'immigrés clandestins de ces arrestations, pour un budget global de 62,5 millions de dollars ! Clairement, l'intervention humaine est moins onéreuse et plus efficace. Pire encore, on apprenait en 2016 que les cartels mexicains pirataient les GPS des drones surveillant la frontière pour la franchir tranquillement. Cette inefficacité est sans doute à l'origine de la volonté de l'ex-président Trump de construire son fameux mur, autre gabegie qui ne connaît guère plus de succès. Concernant l'Europe, Concernant l'Europe, les chiffres montrent l'explosion du budget de l'agence Frontex, de 137 millions d'euros en 2015 à 322 millions d'euros en 2020, selon les chiffres de la Cour des comptes européenne, et une automatisation toujours plus grande de la surveillance des frontières. Parallèlement, le ratio entre le nombre de personnes qui tentent de franchir la Méditerranée et le nombre de celles qui y laissent la vie ne fait qu'augmenter. Cette automatisation de la surveillance aux frontières n'est donc qu'une nouvelle façon pour les autorités européennes d'accentuer le drame qui continue de se jouer en Méditerranée, pour une efficacité qui, finalement, ne profite qu'aux industries de la surveillance. À l'échelle de la France, la problématique est la même : de tels drames humains ont lieu chaque jour dans les Alpes. En plus d'être littéralement inhumaine, la surveillance de la frontière par drones nous semble particulièrement onéreuse et inopportune.

Si l'on voulait respecter les droits à Montgenèvre, il faudrait créer un centre d'accueil, ce qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. On refuse les demandeurs d'asile, on les renvoie en Italie. Je pourrais parler des centres

en parfaite collaboration avec l'Italie. Par ailleurs, nous devons résoudre des problèmes plus profonds, qui sont la conséquence soit des désordres climatiques, soit des désordres économiques, soit des désordres politiques, ce que la France fait très largement puisqu'elle octroie à peu près 30 000 demandes d'asile par an

à l'endroit des réfugiés. Nous sommes des parlementaires et c'est notre travail

extrêmes dans des conditions qui ne sont pas dignes de notre pays et de nos valeurs, mais de surcroît on met les agents des forces de l'ordre en situation de faire des choses que, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ils réprouvent.

A-t-on entendu parler hier de manifestations qui étaient instrumentalisées par des gens qui n'ont qu'une envie : utiliser la liberté et la conviction de ceux qui vont manifester pour détruire ? À Rennes, pendant des mois,

pour assurer la protection des installations militaires et des installations d'importance vitale en définissant les conditions de mise en oeuvre des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord. Il est proposé, à ce titre, d'insérer de nouvelles dispositions dans les première parties du code de la défense pour compléter le régime juridique des installations d'importance vitale et des installations militaires. Ces caméras seront utilisées à des fins de protection des zones militaires et des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale. Dans ces conditions, des garanties propres à ces usages sont définies, tenant notamment à une durée de conservation des enregistrements limitée et à une information générale du public. Les traitements de données mis en oeuvre devront également respecter l'ensemble des garanties de la loi Informatique et libertés, en particulier son article 31. Ces traitements seront ainsi soumis à l'avis préalable de la CNIL. L'acte réglementaire les autorisant déterminera, outre la durée de conservation prévue par les nouveaux articles en cause, les catégories de données traitées, les destinataires de ces données et les modalités d'exercice des droits reconnus aux personnes concernées par ces traitements. Le sous-amendement

Cédric Perrin. En examinant les conditions de fonctionnement et de protection de certaines unités militaires ou de certaines bases militaires, on note cependant qu'une partie des images sont prises par hélicoptère.

d'arrêter un terroriste dangereux s'apprêtant à menacer une installation stratégique à Dunkerque : cette personne avait parcouru des kilomètres le long du littoral. C'est évidemment

le secours d'urgence aux personnes ; la lutte contre les incendies et les accidents.

Le présent amendement est directement inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza et du groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Cet amendement de sagesse vise à instaurer un moratoire interdisant l'usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu'à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales. C'est le choix de plusieurs villes américaines, telles que Portland ou San Francisco.

qui ont été décevants. Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations irrévocables. Elles sont, par définition, uniques et inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue de ces données doit être mise en place. Cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d'éthique et de consentement. La reconnaissance faciale n'est pas, à ce jour, une technologie totalement mûre et possède encore de nombreux défauts techniques, comme cela a été souligné au cours des débats. Il existe, notamment, des biais lorsqu'il s'agit des minorités ethniques, des femmes et des jeunes. Par ailleurs, cette technologie peut engendrer des dérives mettant en danger nos libertés et notre démocratie, comme le démontrent les cas de répression des manifestations à Hong Kong ou la surveillance de la minorité ouïghoure par la Chine. Ce moratoire permettra de prendre le temps nécessaire pour mener et conduire un débat public digne de ce nom. La CNIL ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données le demandent. Un tel moment démocratique permettrait de mieux cerner les attentes de l'ensemble de la société civile en matière de numérique, de coconstruire un cadre normatif et de mener une analyse d'impact rigoureuse sur la reconnaissance faciale. Il s'agit donc tout simplement, comme beaucoup s'accordent à le reconnaître, d'un amendement de bon sens.

et de ses collègues, car nous nourrissons des inquiétudes assez profondes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale.

Malgré tout, il est prématuré de s'engager dans la voie de la reconnaissance faciale. Le ministre nous a assuré hier qu'il n'y aurait pas de reconnaissance faciale, car nous butons parfois sur des questions

deux ans pour éviter que l'on s'engage trop vite et trop mal dans la reconnaissance faciale.

Cet article vise à créer un cadre juridique à l'usage des caméras embarquées dans les véhicules des forces de l'ordre et des services de secours. Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'extension de l'usage des caméras embarquées partout dans l'espace public, et à la surveillance massive et indifférenciée à laquelle cela conduit. Certes, la commission des lois du Sénat a procédé à des modifications de cet article pour y intégrer des garanties complémentaires relatives au traitement des images constituant des données à caractère personnel, bien d'autres points de cet article posent problème. Je pense à l'usage possible de moyens militaires pour surveiller les populations telles que les drones ou encore les hélicoptères équipés non plus d'une « simple caméra », mais d'une optronique », dont la caméra thermique et le zoom surpuissant permettent à la police de filmer, de traquer, d'identifier, de jour comme de nuit, et de retransmettre en direct le flux vidéo, avec une « qualité d'image comparable à celle que le public connaît pour le Tour de France

de la surveillance de manifestations à la surveillance des frontières, ou encore à la surveillance de tous les lieux « ouverts au public ». Je pense enfin au fait que les populations ne soient pas forcément informées de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à cet article.

une pratique qui existe déjà, illégalement, depuis plus de dix ans. Cependant, malgré les modifications introduites par la commission des lois, cet article continue de soulever des interrogations, similaires à celles qui se posent pour l'encadrement des caméras aéroportées prévu à l'article 22 de la proposition de loi. Son champ d'application est trop lâche et ne va pas sans poser de difficultés, notamment lorsque les caméras embarquées sont utilisées dans le cadre de manifestations. Les modalités d'information du public ne sont guère explicitées. Les exceptions posées à l'information du public- l'interdisent et lorsque les objectifs visés s'y opposent -ne semblent pas assez précises et laissent une marge de manoeuvre trop importante aux forces de sécurité. Alors que le respect des libertés fondamentales est en jeu, il n'est pas acceptable de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir le cadre de ce dispositif. Quel est

que soit interdit le traitement des images captées par des caméras embarquées des logiciels de reconnaissance faciale. Je rappelle que la reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. (RGPD) garantit aux citoyennes et aux citoyens européens « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage », selon la définition du profilage inscrite à l'article 4 L'usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l'article 5 du RGPD. Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l'article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique

de vote. Le refus du rapporteur et du ministre me laisse perplexe. Cet amendement est pourtant extrêmement simple : il dit que le traitement par reconnaissance faciale est interdit.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

mais relatif à l'usage des drones. Il s'agit ici, dans le cadre de l'usage des caméras embarquées, de garantir l'information du public par une signalétique spécifique. Autrement dit, lorsque ces caméras sont utilisées et qu'elles filment des citoyens présents dans l'espace public, ceux-ci doivent en être informés par tout moyen. Les exceptions en la matière n'ont pas leur place dans un dispositif aussi problématique que celui qui nous est proposé, avec un éventail d'usages démesuré, puisque notre amendement visant à limiter les finalités aux situations de secours et d'urgence n'a pas été retenu. Vous l'aurez compris, cet amendement revêt

La CNIL n'est pas qu'un organe consultatif. Vous le savez, elle est également chargée d'un travail de terrain. En effet, elle peut notamment missionner un ou plusieurs de ses membres pour procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur tout traitement de données à caractère personnel. Si le recours à la vidéosurveillance est toujours plus important, dans la perspective de sécuriser les locaux et terrains des entreprises et des administrations, il apparaît nécessaire que la CNIL exerce un contrôle actif et efficace concernant le traitement des données qu'impliquent de tels dispositifs. L'objet de cet amendement est donc d'expliciter cette fonction en l'inscrivant parmi l'ensemble des missions dont la CNIL est chargée.

la CNIL a tout à fait la possibilité d'intervenir sur le contrôle des systèmes de vidéoprotection et de tous ceux que nous avons énumérés. Par ailleurs, le président

Vous le savez, ces annonces de la modification à venir du zonage entre police et gendarmerie inquiètent les élus. Même si nous partageons ce constat- oui, la répartition territoriale a, dans certains territoires, perdu de sa pertinence -, une réforme s'impose. Cet amendement ainsi que le suivant visent à introduire davantage de souplesse et d'efficacité. Mais il faut que cette réforme à venir, quelle qu'elle soit, fasse l'objet d'une étroite concertation, en amont et en aval, avec les associations d'élus locaux, afin de réaliser un « délicat travail de dentelle », pour reprendre l'expression de notre collègue Françoise Gatel.

police, alors que de nombreux élus souhaitent basculer en zone gendarmerie. Le sujet est donc sensible dans nos territoires et chez les élus, mais également au sein des forces de sécurité. Même si policiers et gendarmes s'en défendent, chacun dénonce par avance la volonté hégémonique de l'autre. Aujourd'hui le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes de plus de 20 000 habitants relèvent par défaut de la compétence de la police nationale. Nous voulons, par cet amendement, créer une dérogation qui permettrait à la gendarmerie d'assurer la sécurité publique des communes jusqu'à 50 000 habitants.

commission ? Lorsque j'étais député, j'ai défendu auprès de cinq ministres de l'intérieur successifs, sous deux gouvernements d'orientation politique différente, la question du partage entre les zones de police et les zones de gendarmerie. Chaque fois, j'étais accompagné

donc tout à fait fondée et respectueuse des lois de notre République. Vous ne pouvez pas empêcher certains maires, jusqu'au seuil de 50 000 habitants, de vouloir une une représentation plus efficace des forces de gendarmerie ! Tel est le sens de cet amendement, que j'appelle mes collègues à soutenir.

un appel à la souplesse, à l'efficacité, à l'optimisation des échanges et des coopérations territoriales de toutes les forces de sécurité, un appel, enfin, à une intégration plus directe de l'ensemble des acteurs dans ce fameux continuum de sécurité. La clé de répartition arithmétique actuelle entre les forces de gendarmerie nationale et les forces de police nationale ne convainc plus ni les élus ni les forces de police et de gendarmerie. Dans le contexte sanitaire actuel, vous avez pu le constater, les bassins de délinquance évoluent- vous l'avez dit, monsieur le ministre. Les mesures sanitaires ont notamment renforcé les comportements d'occupation du domaine public. Face à ces réalités, les forces de l'ordre sont souvent en nombre insuffisant. insuffisant. La connaissance des problématiques de sécurité en zone périurbaine par les forces de gendarmerie constitue, à mon sens, une indéniable amélioration de la sécurité globale de nombreux territoires. Je citerai ainsi la ville de Carcassonne qui comprend, en plus de sa zone urbaine, cinq hameaux rattachés qui se suivent et dont les populations sont similaires à celles des communes rurales limitrophes. Il convient désormais de dépasser le seul critère démographique de leur répartition sur nos territoires, en tenant compte de leurs besoins ponctuels. Tel est l'objet de cet amendement. Vous me répondrez que la possibilité de renforcer la zone de police nationale par la gendarmerie départementale existe déjà au travers de la coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires (Corat), mise en place en 2011. Ce dispositif prévoit notamment que, dans un cas imprévisible et urgent excédant ses capacités de réponse, une force peut demander le concours de l'autre force. La Corat s'applique pour les communes de toutes tailles, quelle que soit la zone de compétence. Mais nous voulons aller plus loin et prévoir un élément de souplesse si le maire en fait Ainsi, cet amendement prévoit que, dans les communes de moins de 50 000 habitants, à la demande du maire et sous l'autorité du préfet, des brigades mobiles de gendarmerie pourront intervenir en appui ponctuel en zone de police nationale. Les unités de gendarmerie pourront donc venir s'agréger à la police nationale actions dans nos zones urbaines.

Monsieur le ministre, à la fin du mois de novembre 2020, vous avez reconnu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale que la police souffrait de sept péchés capitaux. Vous avez, à cette occasion, fait des propositions de réforme pour répondre,

Vous avez fait des propositions, sans aller très loin dans les préconisations, mais en reconnaissant qu'il existait un problème de transparence et de confiance et qu'il serait peut-être opportun de nommer une personnalité indépendante à la tête Cette réforme de l'IGPN est attendue, parce qu'elle est nécessaire. Les organes actuels de contrôle interne des forces de l'ordre font l'objet de critiques récurrentes en raison de leur manque d'indépendance, qui entretient le soupçon de partialité. L'effet de corps lié à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers et des gendarmes rattachés organiquement au ministère de l'intérieur, les directions générales de la police et de la gendarmerie, crée un sentiment d'entre-soi professionnel et entretient une culture corporatiste. Comprenez bien, monsieur le ministre, que nous ne mettons pas en cause l'action des contrôleurs de l'IGPN en tant que telle. Ces derniers sont redoutés par les fonctionnaires de police, et nous ne disons en aucune façon que l'IGPN est une machine à laver les violences illégitimes. Nous prenons également acte de certaines évolutions réalisées ces dernières années dans le sens de l'ouverture et de la transparence de l'institution- je pense notamment au bilan annuel de l'IGPN présenté à la presse et à la mise en place d'un comité d'orientation du contrôle interne -, mais elles restent insuffisantes, car votre ministère a une capacité de résistance incroyable

Pour y parvenir, il faut séparer la chaîne de contrôle et la chaîne de commandement. À défaut, les forces de l'ordre encourent le risque que les actions qu'elles mènent dans le cadre de leur mission de sécurité publique continuent d'être désavouées et contestées. Cet amendement tend donc à vous inviter, monsieur le ministre, à donner suite à votre engagement de réforme de l'IGPN.

sur l'article. L'article 23 de la proposition de loi prévoit de supprimer les crédits de réduction automatique de peine pour les auteurs d'infractions qui sont commises

qui pose de réels problèmes. D'où la nécessité d'une grande fermeté pénale à l'encontre de ceux qui s'attaquent aux membres des forces de sécurité, des forces de l'ordre et aux élus locaux.

Je l'ai déjà dit, rien dans ce texte n'a été envisagé pour remédier à la culture de l'impunité qui porte atteinte à l'image des forces de l'ordre et contribue à saper le lien de confiance nécessaire entre celles-ci et la population. Alors que nous commençons l'étude du titre IV relatif aux forces de sécurité intérieure, nous nous devons de reconnaître la réalité que vivent certains de nos citoyens au quotidien, malgré le peu d'enquêtes permettant de la documenter, chiffres à l'appui : c'est celle des contrôles au faciès. Selon l'enquête publiée en 2017

observés à plusieurs endroits de Paris, les personnes perçues comme « noires » ou « arabes » ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme « blanches

un dispositif mettant en place, en contrepartie, des garde-fous à l'action parfois abusive des forces de l'ordre. Nous ne pouvons plus faire l'autruche face à ces abus ... La parole

personne est incarcérée dans le cadre d'une condamnation définitive, elle peut bénéficier de deux types de réductions de peine : d'une part, de réductions de peine en fonction, pour le dire de manière simple, du comportement

adapté ou paisible du détenu, sa capacité à s'insérer dans la vie carcérale et sa réinsertion potentielle. C'est par les réductions de peine

recoupe les arguments qui sont les nôtres pour demander la suppression de cet article. Si l'on revient aux dispositions antérieures à 2004,

n° 115. L'article 23 prévoit la suppression du bénéfice des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées à la suite de la commission de certaines infractions graves : meurtres, actes de torture, actes ayant conduit Cette disposition porte atteinte de manière manifeste au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, ainsi qu'au principe d'individualisation de la peine prévu à l'article 132-34 du code pénal.

ou accorder des crédits de réduction des peines, en fonction notamment du comportement de la personne incarcérée. Pour les professionnels de la justice, ces crédits constituent constituent un outil de gestion du bon ordre en détention et permettent, de ce fait, de réduire l'insécurité et l'exposition des surveillants pénitentiaires à des faits de violence. En outre, l'article 707 du code de procédure pénale prévoit que le régime d'exécution des peines est « adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ». Selon les dispositions de ce même article, toute personne incarcérée doit bénéficier d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire. En privant l'administration pénitentiaire et le JAP de leur choix pour accorder ou non ces crédits, l'article 23 rompt avec les objectifs de réinsertion sociale des personnes condamnées et de lutte contre la surpopulation carcérale. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article. La parole

le champ des infractions concernées par la suppression des crédits sur les infractions les plus graves : meurtres, actes de torture, actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ce qui n'était pas le cas dans le texte de l'Assemblée la commission a, par ailleurs, permis d'étendre le champ des personnes au préjudice desquelles ces infractions sont commises pour y inclure les magistrats et les personnes dépositaires de l'autorité publique, notamment les élus locaux,

de votre propos, priver l'administration pénitentiaire de tout outil en matière de crédits de réduction de peine serait irresponsable. Il est vrai que le garde des sceaux nous annonce une réforme en la matière. Nous avons, dans notre amendement, esquissé une première piste pour maintenir un dispositif incitant à la bonne conduite en détention, et donc créer une nouvelle forme de crédits de réduction de peine. Nous avons atteint ce triple objectif dans l'amendement de la commission, raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable aux amendements de suppression. Quel est l'avis

de l'action publique, le président Bas avait lancé une enquête sur la situation des élus. Chacun d'entre nous connaît ou a vécu

que les militaires réquisitionnés sur le territoire national pour garantir la sécurité de tous les Français face aux attaques terroristes bénéficient également des dispositions du nouvel article L. 721-1-2 du code de procédure pénale.

nous obligent. En effet, face à l'augmentation de ces menaces, notre devoir est de protéger l'ensemble de la communauté éducative. En conséquence, cet amendement vise à renforcer la protection des enseignants de l'éducation nationale, mais également de l'enseignement supérieur. Quel est l'avis de la commission ? Je donnerai

nous nous sommes calés sur le dispositif concernant les circonstances aggravantes, qui existe déjà dans la loi. Pour être clair, madame de La Gontrie, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai demandé l'avis éclairé de la Cour de cassation avant de vous présenter l'article. Si je vous le présente comme tel, c'est que j'ai obtenu un avis de « sagesse positive », si j'ose dire.

Je voudrais dire à René-Paul Savary que nous sommes tout à fait sensibles à la démarche qu'il a entreprise avec plusieurs de ses collègues et que la commission des lois intégrera bien cet amendement

sous certaines conditions. La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a élargi les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d'une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d'un numéro d'immatriculation.

les faits commis en raison des fonctions exercées par la personne, même s'ils ne surviennent pas dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. En effet, de nombreux faits divers récents ont malheureusement montré que des délinquants cherchent désormais à identifier les policiers et les gendarmes pour diffuser leurs identités, notamment à travers les réseaux sociaux, dans le but de les agresser, y compris en dehors de leurs heures de service. D'autre part, cet amendement vise à intégrer dans le champ des infractions réprimées les faits commis sur un proche des personnes citées à ces articles en raison des fonctions exercées par ces dernières. constaté à plusieurs reprises la lâcheté des agresseurs qui les pousse désormais à s'en prendre notamment aux conjoints et aux enfants des membres des forces ? M. Karoutchi, comme toujours, a eu une impulsion pertinente puisqu'il propose d'élargir le délit d'embuscade aux actes commis à raison de la qualité de la personne et contre sa famille. Cela va tout à fait dans le sens des propositions de la commission pour plusieurs autres et apporte un complément tout à fait utile au délit d'embuscade. L'avis est donc favorable.

une procédure d'anonymisation des témoignages, afin de protéger les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure. Toutefois, ce dispositif n'est accessible qu'aux témoins dans des procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Cela nous paraît insuffisant et nous demandons un élargissement aux cas d'agression de tout dépositaire de l'autorité publique. permettrait une meilleure répression de ces actes participant largement au climat d'insécurité qui peut parfois régner. Ainsi, cet amendement vise à élargir le principe d'anonymat aux personnes témoins de toutes infractions et agressions envers des dépositaires de l'autorité publique.

tout en l'élargissant aux policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux. Le principe de l'anonymat est déjà inscrit dans la loi, mais uniquement pour les témoins de crimes ou de délits. Cet amendement vise donc à élargir le principe d'anonymat aux personnes témoins de toute infraction d'agressions envers les sapeurs-pompiers, les policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux.

et je comprends, en tant que ministre de l'intérieur et en tant qu'élu, ce que vous souhaitez protéger, puisque, plus qu'avant, les sapeurs-pompiers interviennent dans des conditions extrêmement difficiles et sont agressés. Ils sont manifestement devenus des symboles